la séance est ouverte le parlement est réuni en congrès conformément au décret du président de la république publiée au journal officiel du premier mars deux mille vingt quatre l'ordre du jour appelle le vote sur le projet de loi constitutionnel relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse

les délégations de vote pour le scrutin cesseront d'être enregistrées dans dix minutes le scrutin aura lieu dans salles voisines de l'hémicycle. M.. le président du Sénat,

en venant ouvrir cette séance en remontant avec la solennité qui s'attache à ces lieux à la galerie des bustes d'homme exclusivement

a son époque en effet on ne comptait que treize femmes parmi les députés sept parmi les sénateurs En contemplant aujourd'hui le Parlement réuni en congrès, je constate avec vous que la place des femmes a changé. Parce que la France a changé, même s'il reste beaucoup à faire pour atteindre la parité vraie. Oui, les temps ont changé, l'égalité a progressé, la parole s'est libérée Oui. Hommes et femmes ici réunis, élus de la nation, nous nous à faire franchir à notre pays ensemble un nouveau pas sur le chemin des droits des femmes. Vous comprendrez alors que je sois fier de présider le congrès du Parlement au château de Versailles à cet instant précis où la liberté défendue par Simone Veil va être gravée dans le marbre de notre Constitution. Je suis fier de pouvoir rendre hommage ici à toutes celles qui ont écrit qui ont agi et aussi à celles qui se battent encore. Au quotidien. Près d'ici ou loin de nous, pour que nous escalades mètre par mètre paroi escarpée menant à l'égalité entre la, les femmes et les hommes, car c'est bien une paroi que nous avons à gravir. Paroi dont l'ascension reste longue et laborieuse et trop encore incertaine, et nous savons toutes et tous qu'il suffit d'un instant pour que tout ce que l'on croyait acquis ne le soit plus Alors, oui, nous avons progressé, mais il reste tant à faire sur le terrain de l'égalité et les violences faites aux femmes sont encore, hélas, une tragédie du quotidien. cette nouvelle avancée, il suffisait d'écouter les femmes dans toute leur diversité Quelles que soient leurs conditions sociales, pour se convaincre de la nécessité de s'y atteler Il suffisait de regarder le monde pour se convaincre de l'opportunité de s'y atteler. Les droits des femmes ne sont ils pas les 1ᵉʳˢ à être menacés lorsque le populisme ou l'autoritarisme s'emparent du pouvoir ou que les partisans de l'obscurantisme prétendent nous imposer un ordre moral toujours rétrograde que le monde est secoué de tant de crises notre pays s'attache à renforcer la garantie des droits la france serait elle à contre courant non elle est à l'avant garde elle est à sa place c'est là sa mission et elle est attendue aux femmes de france nous disons que nous ne jamais aux femmes du monde nous disons que nous les soutiendrons et que nous avancerons toujours à leurs côtés je suis fier nous serons fiers demain de ce congrès visant à proclamer que la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse fait désormais partie de notre loi fondamentale. applaudissements Nous sommes dans notre rôle, le Parlement a montré, une fois de plus, que lorsqu'il en a la volonté il sait transcender les clivages politiques pour emprunter le chemin du progrès retenons cette leçon appuyons nous sur la vitalité de la démocratie parlementaire le constituant vient consacrer son œuvre il le fait avec gravité conformément à la seule procédure qui permette de réviser la constitution celle prévue en son article l'heure est venue de nous prononcer l'heure d'exercer ce pouvoir constituant pour nous pour la nation pour toutes les femmes pour toutes nos filles en france et dans le monde je vous remercie

l'acte de procréation est l'acte de liberté par excellence la liberté entre toutes les libertés la plus fondamentale la plus intime de nos libertés

se trouve la mère d'une jeune fille de seize ans dont le crime d'avoir aidé sa fille à avorter après avoir été violée gisele halimi se tient face à une justice d'homme face à une loi écrite par des hommes la liberté de chaque femme

alors que nous vous proposons de l'emprunter un peu plus c'est avec la plus grande humilité que je m'adresse à vous Car oui, Mᵐᵉˢ, et je dis bien, l'homme que je suis ne peut imaginer vraiment la détresse qu'ont pu connaître ces femmes privées de la liberté de disposer de leur corps des décennies durant l'homme que je suis ne peut imaginer vraiment la souffrance ph physique d'alors quand l'avortement était synonyme de clandestinité honteuse, de douleurs innommables et de risques fatal. L'homme que je suis ne peut imaginer vraiment la souffrance morale face au poids d'une société qui préférait taire et condamner. Mais le frère que je suis, le fils que je suis l'ami, que je suis le 1ᵉʳ ministre, que je suis retiendra toute sa vie la fierté d'avoir été à cette tribune en ce jour. Ce jour où sera, je l'espère consacré le combat de femmes et d'hommes de tous bords confondus, de toutes sensibilités confondues, qui font honneur à la nation des droits qu'est la France en ayant rendu possible cet instant. instant. Où nous pouvons ensemble, unis, pleins d'émotions, changer notre droit fondamental, notre loi fondamentale pour yy inscrire la liberté des femmes. Car nous avons une dette morale envers toutes ces femmes et ces femmes qui ont souffert dans leur chair comme dans leur esprit, parfois jusqu'à y perdre la vie. Oui, ces femmes mortes pour avoir voulu être libres, nous hantent, Oui, les aiguilles des faiseuses d'anges nous hantent, Oui, ces échappées clandestines pour avorter à l'étranger. La peur au ventre nous hante. Oui, nous sommes hantés par la souffrance et par la mémoire de tant et tant de femmes quii, des décennies durant, ont souffert de ne pas pouvoir être libres, allant jusqu'à parfois payer du prix de leur vie l'injustice que le législateur exclusivement masculin voulait maintenir sur ma aujourd'hui. ma aujourd'hui. le cours de l'histoire, il est de notre devoir que les consciences qui s'éveillent à présent et celles qui écloront demain ne soient plus hantées par ces souvenirs macabres, mais qu'elle soit plutôt habitée par la fierté que nous leur aurons ainsi léguée, celle d'appartenir à un peuple éminemment libre. conscient que le progrès est un but, que les droits sont moyen et que le corps des femmes n'est rien d'autre que l'empire de leur liberté et de leur libre arbitre et non pas Mᵐᵉˢ et MM.. l'outil d'un projet qui nee serait pas le leur. Alors Mᵐᵉˢ et MM. les parlementaires? Oui. C'est avec à l'esprit le poids de ces siècles de souffrances et d'injustice que je prends la parole devant vous aujourd'hui, que je prends la parole après des mois d'un travail parlementaire transpartisane qui a commencé bien avant ma an pratiquement jour pour jour après l'engagement historique du Président de la République d'inscrire la liberté des femmes à disposer de leur corps dans notre Constitution. Mᵐᵉˢ et MM. les parlementaires, ce vote, c'est donc d'abord un aboutissement, celui d'un long combat. Le 1ᵉʳ combat fut celui du droit de vote et de la citoyenneté, un combat entamé pendant la révolution, incarné par Olympe de Gouges, un combat poursuivi par tant de femmes que le fait par Louise Weiss, qui réinvente la lutte et pense la femme nouvelle par cecil militante infatigable du droit de vote et première femme à entrer au gouvernement avec irène joliot curie et suzanne lacoste en dix neuf cent six à la faveur du front populaire un combat qui ne trouva son issue qu'avec la libération pendant près d'un siècle marianne était une femme mais pas le droit de voter il fallut attendre mille neuf cent pour que l'injustice soit enfin réparée nous sommes au lendemain de la seconde guerre mondiale et enfin les femmes sont vraiment citoyennes enfin elles ont le droit d'être élues et de voter ce pas de géants pour l'égalité nous le devons à l'alliance des gaullistes des communistes des chrétiens démocrates et des socialistes rassemblés autour de l'égalité c'est la démonstration que les plus grands progrès sont le fruit de l'unité, une démonstration que nous sommes à nouveau en mesure de faire aujourd'hui, mais contrairement à l'espoir des réactionnaires, le combat était loin d'être finie car les femmes avaient le droit de vote, mais pas la liberté de disposer de leur corps. Alors il a fallu de la conviction des combats et du temps, trop de temps Les 30 glorieuses sont des années d'accélération. la france se reconstruit se renouvelle se modernise elle oscille entre insouciance et abondance et pourtant les droits des femmes eux n'avancent que lentement le corps des femmes reste un tabou et la loi scélérate de mille neuf cent vingt qui fait de l'avortement un crime passible de la cour d'assises plane au dessus d'elle mais les voix s'élèvent de plus en plus nombreuses

cent soixante douze les procès de bobigny divisent l'opinion gisèle halimi défend les accusés mais prend en réalité la parole pour toutes les femmes avocate des prévenus mais procureurs contre un système qui prétend décider à la place des femmes

souvenons nous des mots qui résonnent et des insultes qui fusent alors dans l'hémicycle à son endroit barbarie, nazisme, génocide, fourré, matoises et tant d'autres, malgré les injures, Simone Veil nee cède pas malgré les insultes et les menaces, Simone Veil ne plie pas. le présentent doit répondre à l'histoire, Alors, Mᵐᵉˢ et MM. les parlementaires, 50 ans plus tard, sous le regard de la famille de Simone Veil, que la force de vos applaudissements pour son combat et pour sa cause tonne plus fort encore que ses insultes et fasse définitivement justice à Simone Veil. Si, peu

Si, peu après sa mort, ont fleuri dans les rues des affiches, des portraits avec ces mots. Merci Simone cela n'a rien d'un hasard le legs est universel son courage est un modèle et il nous inspire encore aujourd'hui collectivement la loi veil marque un tournant elle ouvre la voie enfin mais il restait bien des batailles à emporter nous sommes en mille neuf cent quatre vingt deux et yvetot de de l'interruption de volontaires de grossesse par la sécurité sociale c'est la fin des inégalités sociales pour la liberté du corps

nous vingt deux avec le soutien du président de lamé publique et du gouvernement grâce au travail de parlementaires de divers bords politiques le délai pour recourir à l'i v g est allongé certaines des entraves qui demeuraient sont enfin levées deux mille vingt quatre grâce aux médecins aux associations féministes au planning familial aux é veilleurs de conscience aux élus aux parlementaires aux héritières et héritiers de ces combats passés mais jamais achevé la marche du progrès a fait son office je veux rendre ici hommage à toutes les associations qui ont œuvré et œuvrent encore pour les droits des femmes et, en 1ᵉʳ lieu, pour leur droit à disposer de leur corps. Elles sont les héritières de la voix des femmes de choisir et, bien sûr, du F. Elles portent un combat juste.

Il porte un combat juste et font rayonner chaque jour notre devise républicaine grâce à elles les mentalités ont changé les françaises et les français soutiennent sans équivoque la liberté des femmes à disposer de leur corps car je veux le dire le combat des femmes à ces héroïnes

la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes ne peut pas être la guerre des sexes elle ne doit jamais le devenir c'est un combat pour toute notre société un combat universel un combat pour l'unité républicaine et ce combat nous le gagnerons ensemble femmes et hommes, hommes et femmes, côte à côte et rassemblés et je le dis depuis ce congrès présidé par une femme, la 1ʳᵉ de notre histoire, chère Yaël Braun Pivet, je le dis face à un congrès rassemblant plus de femmes que jamais dans notre histoire. je le dis depuis ce congrès comme chef d'un gouvernement paritaire je le dis comme chef d'un gouvernement déterminé à agir pour la cause de l'égalité sous l'autorité du président de la République qui a décidé de s'engager sur ce chemin nous œuvrons pour faire rimer égalité avec réalité car cette révision s'inscrit dans cette année d'action continue et résolue pour les droits des femmes un combats que le président de la république a porté dès deux mille dix sept alors que ce n'était pas encore une évidence dans le débat politique un combat qu'il a déployé dans tous les champs de la vie de la cité politique économique sociale et sociétale un combat dont il n'a rien cédé et qui est par deux fois la grande cause de ce quinquennat parce que le féminisme est universalisme chemin depuis sept ans aidé par beaucoup d'entre vous, nous avons avancé pour offrir des droits nouveaux, notamment au Mercola, exemple avec le versement automatique des pensions pour la santé des femmes en brisant certains tabous comme l'endométriose ou l'infertilité pour l'égalité au travail dans les carrières professionnelles dans les salaires alors qu'à fonctions égales une femme gagne encore seulement les trois quarts de ce que gagnante un homme c'est pourquoi nous continuerons à agir pour responsabiliser les entreprises pour que les femmes puissent obtenir les mêmes responsabilités pour la mise en place de congés de naissance nous agissons contre toutes les formes de violence et pour que la parole se libère en renforçant notre droit en formant les forces de l'ordre et en protégeant davantage les victimes. Nous sommes encore loin d'être au bout du chemin mais pas à pas l'égalité se rapproche Depuis ce congrès, je le dis aujourd'hui, c'est une étape fondamentale que nous pouvons franchir une étape qui restera dans l'histoire une étape qui doit tout aux précédentes en garantissant la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans notre constitution nous donnons une deuxième victoire à simone veil et à toutes celles qui ont ouvert la voie nous adressons surtout un message à toutes les femmes votre corps vous appartient et personne n'a le droit d'en disposer à votre place mesdames et messieurs les parlementaires le progrès est collectif dit car quand elle se met au service du progrès, rien nee peut vaincre l'unité, le texte que nous examinons aujourd'hui en est la preuve c'est bien du Parlement qu'est venue l'initiative du changement porté par des députés et des sénateurs de la majorité comme des oppositions

je veux saluer ma prédécesseure elisabeth borne pour son engagement je veux saluer l'action déterminante menée par les membres de mon gouvernement, je pense au garde des sceaux Éric Dupond Moretti, infatigable artisan du compromis qui guidé par la force de ses valeurs n'a compté ni son temps ni ses heures pour convaincre pour débattre pour répondre et pour apaiser mais aussi à aurore bergé je sais quel aboutissement représente la réunion de ce congrès pour elle. Je veux remercier ici tous les parlementaires de la majorité comme des oppositions qui ont participé à ce travail. Il est des moments dans la vie d'un pays où l'union ou le collectif ou l'intérêt général doivent extraire des querelles quotidiennes je voudrais Mᵐᵉˢ et MM. que nous un instant au moment que nous vivons, combien de congrès du Parlement firent naître une telle unité, combien de congrès du Parlement, firent naître une telle émotion, combien de congrès du Parlement permirent l'inscription d'un droit essentiel pour les femmes, combien de congrès furent le théâtre. Non de joutes politiques politiciennes mais d'unité de gratitude de l'écriture d'un destin commun. Alors Mᵐᵉˢ et MM. les parlementaires réformer la Constitution est une décision qui nee se prend pas à la légère La dernière réunion de ce congrès pour réviser la Constitution date de 16 ans et il faut toujours avoir la main qui tremble, dès lors que nous touchons à notre norme suprême. Mᵐᵉˢ et MM. les parlementaires, nos libertés fondamentales sont inscrites dans notre constitution, vous déciderez par votre vote d'adopter une disposition qui consacrera comme inaliénable et fondamentale la liberté des femmes à disposer de leur corps c'est le sens même du texte que nous vous proposons aujourd'hui d'adopter c'est le sens même de cet alinéa que nous vous proposons d'ajouter à l'article trente quatre de constitution la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir à une interruption volontaire de grossesse je le sais les débats parlementaires ont soulevé plusieurs interrogations ils ont soulevé aussi des débats auxquels je veux répondre à nouveau. Beaucoup semblent dire que l'ivg ne serait pas menacée comme si, au fond, le sens de l'histoire était inévitable, comme sii, le politique n'avait plus son mot à dire, comme si ce qui était acquis l'était pour toujours je le réfute

et lorsqu'on veut s'en prendre aux libertés d'un peuple, c'est toujours par celle des femmes qu'on commence, pare Simone de Beauvoir, encore une fois, avait raison en une génération en une année, en une semaine. On peut passer du tout au tout, de l'évidence à la lutte par les ans aux américaines, qui doivent se battre pour le droit à l'iv G et de l'insouciance à l'angoisse par ans européenne, hongroise et polonaise pour qui l'interruption Von, volontaire de grossesse n'est plus une liberté consacrée de la liberté à l'oppression en une génération. On a vu les Iraniennes passer du port de la jupe à celui du voile obligatoire. On a vu les Afghanes passer de la liberté d'aller à l'école à l'interdiction de s'instruire. On a vu tant et tant de femmes libres devenir des femmes tuées. oui tuées parce qu'elles refusent de se soumettre n'oublions jamais depuis ces pays. depuis ces pays. les femmes nous adressent un message ne jamais s'endormir, ne jamais baisser la garde, ne jamais subir Alors, Mᵐᵉˢ et MM. les parlementaires gouverner, c'est faire obstacle au tragique de l'histoire, c'est se dresser face aux malheurs du temps présent, bien sûr, mais aussi faire obstacle de toutes nos forces aux tragiques du temps à venir et la politique, c'est faire obstacle à la folie, des hommes, c'est faire obstacle à ce dont on dit jamais ne gouverneront, ne gouverneront jamais, ils n'oseront s'en prendre aux femmes, à nos mères, à nos filles, à noss sœurs peuvent se retrouver à s'exprimer depuis cette tribune sans que personne n'ait jamais cru cela possible, Alors, oui, ce texte est un rempart aux faiseurs de malheur à ceux pour qui tout était mieux avant à ceux qui oublient de dire que, dans cet avant, la femme n'était pas libre à ceux qui sont nostalgiques, d'un temps où la femme ne pouvait pas travailler sans autorisation, d'un homme, d'un temps où la femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sans l'autorisation d'un hommme, d'un temps où la femme ne pouvait pas dépenser son argent, comme ne pouvait pas dépenser son argent comme elle l'entendait d'un temps, Enfin, où les femmes ne pouvaient pas avorter. Inscrire ce droit dans notre constitution, c'est fermer la porte au tragique du passé et à son long cortège de souffrances et de douleurs, c'est empêcher davantage encore les réactionnaires de s'en prendre aux femmes mais légiférer c'est aussi préparer l'avenir cet avenir que l'on aborde bien souvent comme une marche en avant pétri de certitudes et notamment de celles que le progrès serait un aller sans retour jamais jamais nous ne répéterons les erreurs du passé

mesdames et messieurs les parlementaires aujourd'hui la france est pionnière aujourd'hui vous direz la France est fidèle à son héritage, à son identité de nation à nulle autre pareille pays phare de l'humanité Patrie des droits de l'homme et aussi et surtout des droits de la femme aujourd'hui à travers votre vote c'est la nation tout entière qui prend en main son destin et qui ose être le premier peuple au monde à graver dans son texte suprême la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse par ce geste ce n'est pas seulement les femmes que vous honorez

bien sûr beaucoup reste à accomplir mais mesdames et messieurs si vous le décidez notre loi fondamentale sera modifiée pour la première fois depuis seize ans le président de la république présidera une cérémonie de scellement de la loi constitutionnelle pour yy rappeler les racines de cet engagement ainsi consacré. Si vous le décidez, un nouveau saut sera alors apposé sur le livre de notre constitution. Ce saut. Il sera fait de larmes et de sang. il sera fait des larmes qui ont coulé sur les joues des femmes qui ont souffert pour exercer ce droit ou qui ont souffert de nee. pas pouvoir yy accéder. Il sera fait du sang de ce long cortège de femmes qui ont payé de leur souffrance physique et, parfois, de leur vie pour permettre que vous votiez aujourd'hui pour la liberté des femmes, Alors, Mᵐᵉˢ et MM. les parlementaires. Voilà 60 ans, la jeune Annie Ernaux connaissait son événement Combien de générations en ont connu des événements, l'événement c'était un matin froid Un regard goguenard, une réprimande paternaliste, la douleur d'une aiguille, l'argent collecté par tous les moyens, les séquelles, la honte, la clandestinité. Le nouvel événement, c'est aujourd'hui celui qui doit clore une fois pour toutes le monde d'hier notre génération, une génération de femmes, de mères aura dans son calendrier intime et politique dans le décompte de ces années une date marquée à jamais qui ne sera pas leur événement de douleur mais un événement de fierté cet événement c'est ce vote du congrès aujourd'hui et je l'espère le saut du huit mars deux

Merci beaucoup, M.. le 1ᵉʳ ministre, Je vais maintenant donner la parole aux orateurs inscrits pour des explications de vote au nom des groupes de chacune des assemblées. Je rappelle que chaque orateur dispose de 5 min. Le 1ᵉʳ à s'exprimer être le président du groupe Renaissance à l'assemblée nationale, M. Sylvain Maillard. madame la présidente du congrès monsieur le président du c du sénat monsieur le premier ministre mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues Près d'un 1/2 siècle après l'adoption de la loi Veil, nous sommes réunis en congrès afin de consacrer une nouvelle avancée pour les droits des femmes dans notre pays. de la constitutionnalisation de la liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, c'est le principe même du droit des femmes à disposer de leur corps que nous sanctuariser dans la loi fondamentale à la solennité de l'histoire, qui nous saisit en ces lieux. la mémoire s'ajoute la mémoire qui nous oblige de celles et ceux qui se sont tant battus pour que ce jour arrive. C'est dans leur pas nous nous inscrivons aujourd'hui et je suis fier de présider un groupe dont les députés sont si fortement engagés pour cette cause aux côtés du président de la République gouvernement. C'est l'honneur de nos assemblées d'avoir impulsé cette révision constitutionnelle au moyen de plusieurs propositions de lois, à l'instar de celle d'aurore Bergé. Mais aussi grâce au travail de nos commissions des lois et de nos délégations aux droits des femmes. S'il variait dans leurs termes, tous nos textes tendaient un même idéal sanctuariser la possibilité pour chaque femme de choisir Car cette liberté, si chère à tous les Français, n'était pourtant l'objet d'aucune protection supra législative. Or, comment accepter qu'un droit aussi fondamental que celui des citoyennes à disposer de leur corps puisse être l'otage des conjonctures du monde? Parce que nous considérons cette liberté comme fondamentale et intangible aux droits des femmes, notre devoir est de lui conférer une valeur constitutionnelle. Notre Constitution n'est pas seulement la base de notre ordre juridique, c'est le fondement de notre République, le reflet de nos valeurs. La liberté de recourir à l'avortement y a donc Et le Et le terme de garantie assure qu'elle ne puisse être remise en cause, ni en fait, ni en droit, ni aujourd'hui ni demain, par quiconque jamais. Bien sûr, ce vote historique ne marque pas la fin de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais il symbolise ce que le constituant peut accomplir de plus noble. lorsque prévaut l'esprit de consensus Ce combat pour le droit à l'avortement a été et demeure celui des femmes Celles quii ont souffert dans leur chair et dans leur âme de se voir refuser cette liberté, tout autant que celles qui se sont battues pour l'obtenir. Mais cette victoire, aujourd'hui, est celle de toutes les citoyennes et de tous les citoyens. au travers de cette réforme constitutionnelle, La France prouve une nouvelle fois sa vocation universelle en devenant le 1ᵉʳ pays à garantir le recours à l'avortement dans sa loi fondamentale Par ce vote, nous adressons un aux femmes du monde entier. qui voient leurs droits bafoués ou renié pas uniquement dans les régimes autocratiques, mais aussi à noss frontières. Cette consécration est donc celle de la liberté de choisir son destin

ses paroles, les députés Renaissance en auront, les auront et dans le coeur en votant ce jour pour dire à la france et aux françaises votre corps votre choix je vous remercie je vous remercie monsieur le président la parole est à monsieur le président de la commission des lois du sénat pour le groupe les républicains françois noël buffett madame la présidente du congrès monsieur le président du sénat monsieur le premier ministre monsieur le garde des sceaux mes chers collègues nous voici réunis en congrès à l'aube de des cinquante ans de la loi veil sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption de grossesse ce vote est le troisième exprimé par le sénat sur la constitutionnalisation de l'i v g depuis le mois d'octobre deux la chambre haute s'est en effet donné le temps de cheminer sur la question à partir des différentes propositions rédactionnelles qui lui ont été soumises et dont elle a écarté les plus inabouties

comme je cite une équilibre entre la position du sénat et de l'assemblée nationale il est vrai que ce texte reprend des points importants texte que le sénat avait adopté le un er février deux mille vingt trois après qu'il ait été amendé en particulier en plaçant cette inscription à l'article trente quatre de la constitution article qui détermine les compétences du législateur en l'occurrence celle de fixer les conditions et donc les limites du recours à l'i v g et choisissant le terme de liberté préférable à nos yeux à celui de droit qui pourrait ouvrir la voie à un droit opposable le texte innove toutefois en proposant d'inscrire dans la constitution la notion de liberté garantie sur laquelle nous sommes nombreux à avoir exprimé des doutes. Le qualificatif garanti semblant placer la liberté de recourir à l'i V. G et droit constitutionnel. Le Garde des sceaux, se fondant pour l'essentiel sur l'avis rendu par le Conseil d'etat sur ce texte, nous a assurés que tel n'était pas le cas. Le projet de loi constitutionnelle vise la protection de la loi Veil et non son extension. Le terme garantie n'est là que pour guider le législateur dans sa mission, mais ne crée, en aucune manière, de droit opposable. Le but du texte est bien de placer la liberté d'avoir recours à une I V G au même niveau que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine valeur constitutionnelle et la liberté de conscience des professionnels de santé, qui est un principe fondamental, reconnu par les lois de la République. La majorité des membres de notre groupe, Les Républicains du Sénat, a voté ce texte conforme La majorité l'a voté parce qu'il ne change rien à l'équilibre fondamental de la loi Veil, qui repose, d'une part, sur la liberté de la femme qui prévaut pendant 1ʳᵉˢ semaines de la grossesse et ensuite sur la protection de l'enfant à naître qui prévaut sauf bien sûr, avortement thérapeutique pendant la période suivant la grossesse La majorité l'a voté enfin, parce que c'est une consécration qui nee modifie pas la manière de concilier les droits et les libertés constitutionnelles. C'est bien d'ailleurs cette interprétation qui devra guider le juge lorsqu'il aura à connaître de contentieux relatifs à l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Pour conclure, je dirais que nous sommes convaincus que, si des problèmes demeurent, ils ne sont pas à cet instant, à cet instant. D'ordre juridique, ils sont avant tout aussi d'ordre matériel. Le groupe Les Républicains s'inquiète depuis longtemps des difficultés d'accès à l'interruption volontaire de grossesse. La constitutionnalisation ne changera malheureusement rien aux difficultés rencontrées aujourd'hui par de nombreuses femmes. Je voudrais sur ce point citer Mme Marie Mercier, notre collègue sénatrice, qui a parlé d'un nouveau départ à l'occasion des débats pour faciliter l'accès à cette liberté et le suivi des femmes. Elle marquera seulement, mais c'est déjà un pas extrêmement important. Un attachement renforcé à une liberté des femmes, affirmée voici déjà presque 50 ans, mais en aucun cas elle ne doit pour autant conduire à imposer une rupture de l'équilibre fragile qui a permis à notre société française la pleine acceptation de cette liberté.

que notre groupe votera majoritairement pour la constitutionnalisation une partie de celui ci s'abstiendra et d'autres voteront contre monsieur le président la parole est à madame la vice présidente hélène pour l'assemblée nationale et le groupe rassemblement national merci madame la présidente du congrès monsieur le le président du sénat monsieur le premier ministre mesdames et messieurs les ministres chers collègues parlementaires étonnante solennité que celle de cette journée du quatre mars deux mille vingt quatre ou dans une france par ailleurs en proie à des tensions d'une ampleur inouïe les deux assemblées de la république se réunissent en congrès afin de voter quarante neuf ans après la dépénalisation de l'l'avortement l'inscription de ce droit dans notre constitution présentée et adoptée pour offrir aux femmes un cadre légal sûr afin de mettre fin à l'horreur de l'avortement clandestin la loi veil pour révolutionnaire qu'elle était porte en elle la marque de la vive conscience de son auteur qu'elle ne régissait pas un acte médical ainsi ainsi prévoyait elle dans son article premier aujourd'hui codifié que je cite la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie la loi mille neuf cent soixante quinze s'est voulue et demeure un texte d'équilibre et de responsabilité si dans les décennies qui suivirent le cadre légal posé weill fut réformé à de nombreuses reprises ce fut toujours dans le sens d'un assouplissement des conditions d'accès à l'ivg

c'est paradoxalement l'idée inverse qui s'est installée celle que le droit à l'i v g était en danger qu'il était urgent de le constitutionnaliser pour le protéger d'une supposée future majorité qui cherche fin ce qui n'est pourtant le cas d'aucune formation politique actuelle de loi constitutionnelle les dépôts de propositions de loi constitutionnelle se sont succédé et qu'une première navette parlementaire a permis d'aboutir à un texte repris à quelques mots près par le projet gouvernemental que nous votons à travers à travers ce texte le gouvernement a heureusement fait le choix de la prudence en inscrivant l'i v g a l'article trente quatre de la constitution il confirme la pleine autorité du législateur pour en fixer les conditions dans la limite d'une loi qui interdirait totalement l'i v g ou priverait à l'égalité de toute effectivité ainsi la lettre constitutionnelle laisse au législateur le soin de trancher la question si lourde de conséquences du délai de plus la notion de liberté garantie à à distinguer de celle de droit opposable n'est pas de nature à remettre en question l'objection de conscience des praticiens nécessaire corollaire de la singularité de cet acte médical constamment reconnue par la loi depuis mille neuf cent soixante quinze dont nous regrettons toutefois l'absence de mention dans ce texte qui aurait permis une plus grande clarté ainsi si l'opportunité de cette réforme interrogea le travail parlementaire a de toute évidence abouti à un texte qui laisse peu de place à la créativité interprétative du Conseil constitutionnel. Aussi, si les députés de mon groupe voteront chacun selon leurs légitimes convictions, nous approuveront ce texte rappelant ainsi clairement à qui de bonne foi craindrait le contraire qu'en aucun cas il ne serait envisageable de revenir sur cette liberté. Gardons nous néanmoins de tout triomphalisme déplacé à propos de ce vote que certains voudraient historique en consacrant en grandes cérémonies un droit que personne ne menaçait la majorité peut gêner il y a deux ans des lies à la tête du Parlement européen une femme au positionnement résolument anti V G s'achète à peu de frais Une image d'épinal pour sa postérité pendant que l'ethnie pèse dans un. le féminisme flamboyant se change subitement en mutisme dès qu'il est question des menaces réelles pour les droits des femmes, à commencer par l'islamisme, sauf celle d'un grand foire institutionnel. En réalité, en réalité au lendemain de ce congrès rien n'aura changé pour les femmes et les chiffres de l'avortement resteront le reflet de tous les progrès sociaux que vous n'avez pas su réaliser

personne n'est ici garant de sa mémoire personne que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. parmi ces actes plus nombreux que jamais et qu'aucune norme ne rendront jamais anodin combien auraient pu être évités par une meilleure instruction sur la fécondité et la contraception, un meilleur accompagnement des femmes, notamment économiques, quii permettrait à toutes celles qui le veulent de mener leur à terme et d'élever leurs enfants dans des conditions dignes. Toutes les statistiques le démontrent, la fréquence de l'avortement et les traitement corrélé à la précarité Aussi, mes chers collègues, que chacun de nous soit lucide sur ce fait tant que nous échouerons collectivement à de répondre à cet immense défi, la liberté que nous consacrons aujourd'hui ne sera jamais qu'une 1/2 liberté. Je vous remercie, La parole est à présent Mᵐᵉ Laurence Rossignol, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat

Quelle fierté, oui, c'est une victoire. n'ayons pas peur des mots

c'est fini arrêtez de vous agiter les français ont choisi nous continuerons Notre vote va également réparer quelques pages noires de l'histoire nous allons réhabiliter toutes les femmes poursuivies condamnées et même guillotinées pour avoir procédé ou subi des avortements

Quelle fierté ces dizaines de messages reçus la semaine dernière du Brésil, des États Unis, de France, de Hongrie, bravo et merci, nous disait elle toutes

Cette sécurisation de l'i V G dans la Constitution, nous la devons d'abord à la société civile citoyenne et militante, nous la devons aux Français et aux Français quii de sondage en sondage ont toujours dit clairement qu'ils voulaient cette réforme, nous la devons aux féministes, ces dizaines de milliers de femmes connues ou anonymes, quii ont maintenu sur le Parlement et l'exécutif, une pression constante jusqu'à ce que le Président de la République prenne le relais. prenne le relais. Qu'allons nous faire? maintenant? Les féministes vont elles enfin partir en vacances? nee? rêvez pas? Ehh bien, non, nous allons continuer, nous allons d'abord continuer pour toutes les femmes, ces centaines de millions dans le monde qui n'ont pas notre chance et n'ont pas accès à l'avortement, nous allons continuer pour celles qui résistent à Trump, à Orban, à Miley, à Poutine, à Mais sans

Mais sans oublier, bien sûr, dans cette liste, celle qui résiste aux mollahs et aux dictateurs théocratiques.

le droit de disposer de son corps de choisir et non de subir sa maternité est la condition de l'émancipation des femmes, mais ce n'est pas un aboutissement Tant que les viols, les féminicides, les inégalités salariales se poursuivront, nous continuerons, tant que le sexisme d'atmosphère perdurera, nous continuerons enfin, chers collègues. Avec notre vote, nous allons faire du bien au pays. À nos concitoyens, ils seront fiers, d'abord fiers d'eux mêmes et, je l'espère, fiers de nous. Aujourd'hui, la France retrouve le fil de son histoire, l'histoire du pays des droits humains et le pays qui donne du courage partout et ceux qui luttent la France qui est là, au congrès, aujourd'hui, c'est la France qui rayonne, pas celle qui s'enferme, ou se recroqueville, Notre vote est un formidable antidote au déclinisme. Il ravive les couleurs de notre devise liberté, égalité, fraternité. vous m'autorisez à ajouter sororité. Vous l'avez compris, le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat votera la constitutionnalisation de l'ivg vive le féminisme Vi de la République et vive de la France.

madame la présidente du congrès monsieur le président du sénat monsieur le premier ministre mesdames et messieurs les ministres collègues aujourd'hui au monde aujourd'hui en entrant dans l'histoire des nations pionnières des droits des femmes la france sonore treize la nouvelle zélande devenait le premier pays au monde à reconnaître le droit de vote des femmes en mille neuf cent six c'est la finlande où les femmes obtenaient les premières le droit d'être élus au parlement quatre le la france renoue avec sa vocation de phare des droits humains quand il yy a un peu plus de deux siècles sa révolution a inspiré le monde aujourd'hui c'est la france qui va pour la première fois consacrer le droit à l'avortement dans la constitution aujourd'hui notre est une promesse faite à l'avenir, une protection que nous devons à la moitié de l'humanité, pour laquelle la nuit n'a que trop duré. C'est avec émotion et fierté que je me tiens devant vous alors que j'ai eu l'honneur d'initier le premier vote à l'assemblée nationale pour constitutionnaliser l'ivg que le mouvement famille dépend depuis deux je salue mélanie vogel qui a ouvert la voie au sénat et toutes les parlementaires engagés dans ce combat ce moment historique a été arraché par une victoire parlementaire, mais ce sont surtout des décennies de combats de militantes, de collectifs et d'associations comme le planning familial que faisons entrer aujourd'hui dans notre norme suprême cette victoire nous la voulons comme un hommage à celles qui ont tracé le chemin de madeleine pelletier infatigable militante pour les droits absolus des femmes à disposer de leur corps dès mille neuf cent onze morte internée d'office dans un asile pour avoir aidé une jeune femme violée à avorter

cette victoire nous l'arrachera en mémoire de celle dont on a retenu le nom mais aussi de toutes les anonymes qui sont restés dans l'oubli. nous l'arracher avec et pour celles qui continuent de se battre aujourd'hui et savent comment ce droit est fragile cette victoire. nous la voulons fondatrice, annonciatrice d'une série de victoires futures ici et ailleurs et alors que nous voterons ce texte. Les Polonaises ont regagné le droit à la contraception d'urgence. notre vote aujourd'hui. Dans le sens d'une reconnaissance, celle de l'avortement comme droit fondamental humain, car il pèse toujours sur les droits des femmes, la menace d'une régression, car le droit à l'avortement figure toujours en 1ᵉʳ sur la liste des conquêtes à abattre l'extrême droite comme en argentine où le nouveau président ravier mile a déjà annoncé avoir pour priorité d'abroger l'avortement comme en pologne où six femmes sont mortes la quasi interdiction de l'avortement

n'en déplaise aux réactionnaires notre corps n'a pas de mission qui lui préexistent le sens d'une vie, est toujours celui que l'on décide d'écrire, c'est l'histoire du féminisme, est celle de l'émancipation, d'une destinée utile unique. l'histoire du féminisme et l'histoire de ce devenir indéterminée où chacune se fait sujet de son propre existence. Pour cela le droit à l'avortement est au carrefour de l'intime et du politique la condition fondamentale dont dépend toutes les libertés la la condition de notre égalité réelle à construire avec les hommes nous continuerons de nous battre pour abroger la double clause de conscience pour que les sages femmes puissent réellement réaliser des I V G instrumentales l'avons nous gagné aujourd'hui pour que l'accès à l'avortement soit effectif alors qu'une femme sur quatre doit changer de département pour pouvoir mettre fin à une grossesse non désirée, Nous continuerons de nous battre pour inscrire le droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'union européenne mais aujourd'hui, Nous célébrons une victoire historique. Notre vote est une promesse faite à l'avenir plus jamais, nos enfants, petits enfants et arrière petits enfants n'auront à revivre les supplices qui ont précédées. Notre vote est une promesse aussi pour pour toutes les femmes qui luttent partout dans le monde. pour le droit à disposer de leur corps, en Argentine, aux États Unis, en Andorre, en Italie, en Hongrie et en Pologne comme en écho Ce vote Aujourd'hui, dit, votre lutte est la nôtre, cette victoire est la vôtre. J'ignore où se livrera le combat entre le vieux monde et le nouveau mais, peu importe, j'y serai à notre manière, nous yy sommes. Aujourd'hui, la France fait son entrée dans le siècle des droits des femmes dès aujourd'hui que toute femme choisisse elle même sa destinée, merci madame la présidente

madame la présidente du congrès monsieur le président du sénat mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues

elle qui disait la femme a le droit de monter sur l'échafaud elle doit avoir également celui de montée à la tribune et aujourd'hui nous y sommes la peine de mort est abolie, les femmes sont à la tribune Président, au Congrès, Mᵐᵉ la Présidente, et ensemble, nous allons écrire l'histoire en inscrivant le droit à l'avortement dans notre Constitution. ici réunis, nous sommes les héritiers de l'âme de Gouge, mais aussi de Simone Veil, de Gisèle Lucien Neuwirth et de toutes celles et ceux qui ont compris que l'universalité se conjugue au masculin comme au féminin. Mesurons le chemin parcouru par notre société il y a 50 ans l'avortement était un crime pour la loi. et une honte pour l'opinion, l'opinion, yy sont aujourd'hui farouchement attachés. Ce chemin parcouru par des mouvements féministes et humanistes qui se sont succédé C'est le nôtre, aujourd'hui parlementaire de tout bord. Rendons en particulier hommage aux deux rapporteurs, Guillaume Gouffier Valent pour l'assemblée nationale Canaille pour le Sénat, partisan de cette réussite. Nous le Nous le savons, certains d'entre vous n'ont pas favorables à cette constitutionnalisation. Estimant que ce droit n'est pas actuellement menacé Merci toutefois d'avoir contribué à ouvrir le débat et à faire de ce moment un grand temps démocratique, un moment dont notre Parlement sort grandi, un moment dont notre nation sort renforcée, et je le crois plus un. Remercions aussi ceux qui ont su que ce soit nous qui sommes leurs collègues, mais aussi Ch, chez eux, leur mère, leur fille, leur femme, leur sœur, leur compagne. Merci également à tous ceux qui, en fin de compte, ont confiance, ont su mettre de côté leurs réserves et leurs doutes pour voter à nos côtés. c'est sans doute aussi ça le courage de surpasser des clivages politiques pour être attentif aux demandes d'un peuple et être au rendez vous de son histoire. Mais c'est parce que ce droit a dû être conquis avant d'être acquis, parce que nous nous remémorons les souffrances de nos mères et de nos grands mères parce que nous saluons leur combat mais nous refusons de le réitérer que nous nous sommes engagés dans cette protection Et au delà du long combat des associations, des militantes, des hommes et des femmes de nos deux assemblées, ce qui nous rassemble, c'est une certaine idée. cette idée que la patrie des droits de l'homme, celle qui a tant brillé par ses positions courageuses, ses novatrices. est aussi celle du droit des femmes Alors oui, cette constitutionnalisation pourrait ne jamais être qu'un symbole, mais quel symbole et comme j'aimerais donner raison à ceux qui le pensent, comme j'aimerais me tromper, comme j'aimerais que jamais cette révision constitutionnelle nee serve, ou que, par sa seule existence, elle dissuade demain toute menace contre l'avortement. Alors, pour le symbole ou pour la protection, offrons à cette liberté ce que notre République a de plus fort notre Constitution. écrivons dans notre Constitution que jamais la liberté des femmes à disposer de leur corps ne doit souffrir d'entraves. Mes chers collègues, nous allons écrire l'histoire et alors que nous nous séparerons et que la vie politique reprendra ses droits. Je souhaite que cette journée nee soit pas une fin mais une promesse. Une promesse que nous faisons aux femmes de ce pays qui auront un jour à recourir à l'i nous saurons vous accompagner avec dignité. Une promesse de nous montrer collectivement à la hauteur des aspirations françaises, des aspirations profondes d'égalité et de liberté des Françaises. Faisons de la France un modèle, car si voter ce texte est un aboutissement pour nous, pour les femmes du monde entier, c'est un espoir, beaucoup reste à faire, c'est demain que tout commence. Je vous remercie La parole est à M. le président Olivier Marleix, pour le groupe Les Républicains à l'assemblée nationale.

en votant aujourd'hui les députés les Républicains s'inscriront dans la filiation historique de la droite en faveur de la liberté des femmes rappelons le c'est le général de gaulle quii mille neuf cent quarante quatre c'est la droite avec lucien levert qui donna la légalisation de la contraception et c'est le président giscard d'estaing qui a eu le courage de porter la légalisation de l'ivg simone veil bénéficiant aussi de l'engagement sans faille du premier ministre jacques chirac L'ivg était il aujourd'hui en danger dans notre pays au point qu'il faille l'inscrire dans la Constitution, nous pouvions en débattre aucun parlementaire n'a jamais eu depuis 50 la moindre initiative visant à restreindre l'accès à l'i v g aucun parlementaire n'aurait j'en suis évidemment absolument convaincu quelles que soient ses convictions le projet fou de renvoyer l'ivg à la clandestinité tragique d'avant soixante quinze qui coûta la vie à tant de femmes mais sans parler des états unis autour de nous au sein même de l'union européenne il y a la restriction du droit à l'avortement en pologne et en hongrie ces menaces ne peuvent pas nous laisser indifférents, et même si ce risque est lointain, nous acceptons de le voir en face et c'est la raison pour laquelle la grande majorité des députés des Républicains voteront pour cette modification de la Constitution. Il est aussi un autre risque plus tangible celui de défaire le six sage équilibre voulu par simone veil en faisant désormais de l'i v g un droit absolu qui écraserait

Or, le gouvernement a fait le choix, avec cette liberté garantie, d'une rédaction a fait planer les incertitudes qui ont été au cœur de nos débats. Est ce que cette liberté garantie qui n'est rien d'autre qu'un droit comme l'a rappelé le garde des sceaux ne viendra pas rompre l'équilibre et la tempérance voulue par pour Simone Veil, la protection de l'enfant à naître en effet Simone Veil avait pris soin d'écrire un article 1ᵉʳ qui précisait je cite La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité ou selon les conditions définies définies par la présente loi devenir ce principe puisqu'il ne sera pas lui inscrit dans le texte constitutionnel, concrètement l'inscription du droit à l'I. V. G dans la constitution ouvre t elle une brèche exploitable pour ceux qui voient dans la limite de 14 semaines une entrave insupportable et un droit fondamental? alors nous avons parfaitement entendu les les assurances répétées du garde des sceaux qui s'est d'ailleurs beaucoup plaint de devoir autant rabâcher durant nos débats la réponse c'est que le principe du respect de l'être humain dès le commencement de la vie ce principe posé par simone veil à l'article premier de la loi de soixante quinze s'intègrent déjà au principe de humaine auquel le conseil castiel a donné une valeur constitutionnelle au terme de nos débats et grâce aux répétitions du garde des sceaux il est donc clair et manifeste que la volonté du constituant que, demain comme hier, le législateur continue de concilier un droit et un principe qui ont tous deux une même valeur constitutionnelle même si l'un est écrit et l'autre pas. Nous prenons acte aussi des garanties apportées sur le maintien de la clause de confiance des soignants le choix d'une rédaction moins ambiguë, comme celle proposée par notre collègue Philippe Bas au Sénat aurait peut être permis une adoption encore plus consensuelle et plus large, quoi qu'il en soit. Ce vote, nous le devons à la liberté des femmes. La parole est à présent, M.. le président François Patria, pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendant du Sénat.

nous rappelle qu'ils sont rares les moments d'unité en politique et c'est donc avec nous aussi, avec fierté, que nous pourrons voter avec beaucoup d'émotions loi et inscrit dans la Constitution le droit à l'i V G. Nulle part les droits des femmes ne sont définitivement acquis, la liberté et l'égalité des femmes ne sont pas des droits acquis, ce sont des combats et qu'il faut sans cesse mener le 8 mars Journée internationale de la lutte des droits des femmes est l'occasion de rappeler combien ce combat quotidien et universel mérite d'être poursuivis la liberté de recourir à l'i V G est souvent ciblée L'actualité internationale nous rappelle que cette liberté fondamentale une fragilité inouïe alors même que le contrôle de la procréation entre les mains. des femmes est la 1ʳᵉ marche V. l'égalité écrivait à François Héritier. Beaucoup de proposs d'une haute tenue, que j'ai saluée et que j'ai applaudi ont déjà été tenus même si des répétitions doivent être dites je voudrais moi aussi insister sur quelques points hors ce combat pour l'égalité des femmes n'avance pas même sous les vents déchaînés des fondamentalistes religieux et des populistes

états n'autorisent plus du tout et cinq autres en restreignent l'usage la contagion se propage partout les opposants à l'avortement se réveillent encouragés par le contexte américain et l'inquiétante des extrêmes droites conservatrices réaction chaînes la porte de la régression s'est ouverte aussi à l'europe cela a déjà été cité les menaces de la liberté des femmes prennent de l'ampleur surtout dans les pays de l'est particulièrement en pologne ce pays qui avait interdit l'avortement en quatre vingt treize sauf exception là encore restreint en deux mille vingt même s'il a depuis un peu reculé le gouvernement de viktor orban mène une politique nataliste sans fard et la constitution a été modifiée en deux mille onze pour inclure la protection de la vie du fœtus dans ce prolongement vingt huit hôpitaux ont alors d'emblée déclaré ne plus vouloir effectuer d'i pas moins de onze propositions de loi visant à limiter l'accès à l'avortement ont été déposés en deux mille dix huit un schéma similaire a été observé en lituanie où des offensives ont rythmé la vie du parlement dix huit un projet proposant même d'aligner la législation sur celle de la pologne s'ajoutent à ces reculs les résistances dans les pays où les droits des femmes semblent les mieux reconnus à défaut de pouvoir interdire l'avortement des pays organisent son impossibilité faute de médecins acceptant de le pratiquer faute de prise en charge des patientes faute de place avec la réduction des centres d'v d'autres pays certains pays ou si la loi dit le médecin dit en croatie soixante des médecins sont objecteurs de conscience dans certaines régions d'italie ce sont jusqu'à soixante dix des médecins qui recouvrent à la clause de conscience la situation est particulièrement dramatique à naples où seul un quart des établissements médicaux pratiquent les v g les g s'avèrent difficiles aussi en bavière avec moins d'une dizaine de cabinets accessibles en deux mille vingt et un même les pays qui se croient à l'abri font l'objet d'offensives les courants anti choix nee renoncent jamais et font preuve de beaucoup d'imagination le dge trr me droite européenne est à la manœuvre et la bataille fait rage n'ayons pas de croire que ce vent mauvais s'arrêtera de souffler à nos frontières ce serait une faute morale et politique, une faute vis à vis des Françaises et des Français qui soutiennent l'inscription de l'ivg dans la Constitution dans dans une très grande majorité et je tiens, ici à saluer Le combat magnifique et sincère, rappelé par beaucoup d'entre vous courageux et sans faille des associations féministes, de tant de femmes célèbres et anonymes, se sont battues pour faire respecter cette liberté pour les femmes de choisir leur vie leur combat est plus que jamais d'actualité la chaîne de désinformations s'ensevelir mer que l'avortement était la première cause de mortalité dans le monde les opposants à l'avortement n'ont jamais désarmé depuis un demi siècle parce que fondamentalement c'est de la liberté et l'égalité des femmes qu'ils refusent au nom d'un modèle social rétrograde vient à la france qui reste aux yeux du monde le symbole de la liberté et de l'égalité d'en réaffirmer solennellement les principes et de garantir dans le texte sacré la constitution cette liberté fondamentale pour la femme, de choisir sa maternité. Oui, il faut protéger les femmes françaises des déséquilibres politiques, ce partout où les extrêmes avancent et les droits régressent. chers collègues, la France devient le 1ᵉʳ pays au monde à rendre irréversible la liberté des femmes, à recourir à l'ivg et à garantir la marche V. L'égalité, c'est un signal universel, pays des lumières, la France peut s'honorer d'être aujourd'hui le phare pour éclairer la les voies de l'avenir et l'immense espoir de toutes les femmes d'europe et du monde. Att avancée, mes chers collègues répondent à de Simone Veil, que tous avaient citée ici nee. Soyons pas de ceux ou de celles qui redoutent l'avenir je vous remercie La parole est à présent à Mme Geneviève Darius, pour le groupe démocrate de l'assemblée nationale.

c'est avec une vive émotion que je m'exprime au nom du groupe démocrate moderne et indépendant devant ce congrès réuni aujourd'hui pour écrire une nouvelle page des droits des femmes

mais il faisait déjà écho à de nombreux drames proches ou lointains quelle force quelle abnégation quel courage ce discours puissant d'âpres débats conclut par des votes favorables à de l'assemblée nationale et au Sénat, c'est diffusé dans tout le pays jusqu'au plus profond de nos campagnes, et cela sans l'aide d'aucun réseau social ni de chaînes d'information continue, tant l'enjeu était immense. Quelle victoire pour toutes les femmes qui ont porté haut le combat de l'autorisation de l'ivg en france après celui de la légalisation de la contraception

qui ne pouvaient s'exprimer qu'en comité restreint je pense à toutes ces femmes qui subissaient en silence ce sont nos mères, nos tantes, nos grand'mères, ce sont elles que j'ai d'abord connues et je peux vous dire que je pense à elles aujourd'hui les mots de Simone Veil. Sonnent encore. Aucune femme nee recourt de gaieté de cœur à l'avortement. car oui recourir à l'avortement aujourd'hui encore est un choix intime et toujours très douloureux

alors nous avons cru que ce combat était gagné en occident que ce droit à la dignité des femmes était conquis définitivement et que les progrès sociétaux continuerait d'avancer inéluctablement pouvait on imaginer en ce début du vingt et unième siècle que de nombreuses démocraties menaceraient cette liberté la pologne et la hongrie n'ont pas hésité pouvait on imaginer que les états unis révoquerai le droit fédéral à l'avortement au moins quatorze états n'ont pas hésité ce recul des droits des femmes ces mouvements de défiance sont inquiétants et inacceptables la dignité des femmes n'est pas négociable c'est un combat qu'il nous faut mener quotidiennement sans relâche. Inscrire la liberté garantie pour toute femme de recourir à l'ivg dans notre constitution n'est ni inutile ni superflue c'est une volonté forte et exigeante pour le présent et pour le futur c'est protéger ce droit et affirmer notre indéfectible attachement aux droits des femmes et des hommes en mille neuf cent soixante quatorze valéry giscard d'estaing s'est engagée à légaliser l'interruption volontaire de grossesse il a confié à simone veil sa ministre de la santé sous jacques chirac son premier ministre le soin d'écrire et de porter cette loi devant parlement ils sont entrés dans l'histoire de l'évolution eton des droits des femmes aujourd'hui cinquante ans plus tard nous sommes réunis ausi en congrès

les parlementaires femmes et hommes de tous bords politiques ont œuvré avec le garde des sceaux pour trouver les solutions d'un vote large dans les deux assemblées Permettez moi d'avoir une attention particulière pour Erwan Balan qui, au nom de notre groupe, a travaillé avec acharnement pour que ce projet de loi aboutisse. Alors oui, nous devons être aujourd'hui au rendez vous de l'histoire de notre pays et, par ce vote, en écrire collectivement une nouvelle page les femmes de France et ainsi faire de la France une pionnière la 1ʳᵉ a gravé ce droit fondamental dans le marbre de la Constitution un message fort pour toutes les femmes du monde. Je vous remercie. La parole est à M.. le président Claude Malu, pour le groupe Les Indépendants République et Territoires du Sénat madame madame la présidente du congrès monsieur le président du c du sénat monsieur le premier ministre mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues je ne vais pas vous parler aujourd'hui de droit constitutionnel je voudrais si vous me le permettez vous raconter une histoire une histoire que je n'ai jamais racontée cinq ans j'étais coopérant médecin chef d'un petit hôpital dans un coin perdu dans un pays du sud l'hôpital est un bien grand mot car les maigres équipements dont il disposait à peine fait classer chez nous comme un dispensaire quant à médecin chef titre ronflant puisque en fait j'étais tout simplement le seul médecin dans cette circonscription de cinquante mille âmes avec une équipe d'infirmiers formidables habitué à travailler seul pendant le semestre ou l'année qui séparait habituellement le départ d'un coopérant français de l'arrivée de son successeur un jour après avoir entendu du remue ménage dans le couloir j'ai vu surgir dans mon bureau une jeune femme dix sept dix huit ans peut être dont je me rappellerai toujours le visage les joues rondes d'une adolescente toute rouge et inondée de larmes essoufflé une expression mêlée de terreur dans le regard Les cheveux décoiffés, les vêtements de travers, comme si elle venait de se débattre. Les bras maintenus par deux gendarmes qui l'encadrent et la poussaient dans la pièce sans ménagement. Le matin même, un voisin, intrigué par le manège de chiens errants qui s'acharnaient à gratter la terre près de sa maison, s'était approché et avait découvert le cadavre d'un nouveau né à peine enfoui dans le sol. L'enquête n'avait pas été bien difficile et l'on me demandait désormais d'examiner la suspecte pour savoir si elle venait ou non d'accoucher j'étais pétrifié Il s'agissait d'un infanticide, bien sûr et la loi Mee commandait de m'exécuter, mais je savais aussi parfaitement pourquoi cette jeune femme était là dans un pays comme tant d'autres où fille mère, c'était le mot de l'époque signifiait bannissement social et pour la famille où où l'avortement était interdit et sévèrement puni Et d'ailleurs comment cette quasi enfant aurait elle pu se confier à quiconque pour trouver une faiseuse d'anges. J'imaginais sa vie au cours des derniers mois. Engrossés par un séducteur de barrières peut être, comme souvent par un parent, découvrant d'abord effrayé son retard de règle puis voyant son ventre s'arrondir et masquant sa grossesse avec de plus en plus de mal accouchant seul en se cachant enterrant maladroitement l'enfant sur place folle de douleur et de culpabilité, puis rentrant chez elle et lavant ses vêtements dans la terreur d'être découverte. Et puis les chiens, le voisin, découvrant le cadavre, les gendarmes et, désormais, le médecin, moi Je suis resté longtemps assis, le visage caché dans les mains cherchant désespérément comment éviter l'inévitable seules la jeune femme et l'infirmière étaient restées près de moi parlant ensemble dans leur langue que je ne comprenais pas au bout d'un moment sollicité par les gendarmes qui s'impatientaient l'infirmier major est entré dans la pièce suivi par l'un d'eux surpris par la scène pressé par le brigadier et n'ayant manifestement pas la même vision du monde que moi, ni les mêmes scrupules avant que j'aie pu faire un geste s'il s'est approché de la jeune femme, a abaissé son mamelon, d'où a giclé le lait qui confirmait le diagnostic et les soupçons, je revois encore cette adolescente. redoublant de pleurs, ressortir accablée entre ces deux gardes Je repense souvent à elle et à ces yeux d'animal traqué et moi me demandant combien d'années de prison pour un infanticide et surtout, combien d'années de culpabilité peut être toute une vie pour avoir tué son enfant. Des je pourrais vous en raconter d'autres si nous en avions le temps des avortements clandestins qui se terminent mal, des condamnations, des stérilité définitives. nous, aujourd'hui, ces histoires n'existent pluss depuis la loi veil et les interventions de ceux qui m'ont précédé ont porté notamment sur le fait de savoir si la liberté de l'i v g risque un jour d'être remise en question. J'ai voulu aborder un autre versant de ce débat et vous dire que 40 au moins des femmes dans le monde vivent dans des pays où des drames, tels que celui que je vous ai retracés, continuent parce que rien n'a changé. En étant le 1ᵉʳ pays au monde à garantir cette liberté nous allons susciter là où nous sommes encore sinon un exemple, du moins une référence des débats, des prises de positions, des avancées, J'espère qui rapprocheront le jour où, comme ici, les femmes seront libérées de la peur de la culpabilité et de l'impuissance à maîtriser leur destin. Au moment de voter mercredi dernier au Sénat, j'ai revu une fois de plus le visage de cette jeune femme dont la vie et celle de son bébé ont été anéanties et je le reverrai tout à l'heure lorsque j'irai voter à nouveau en espérant que mon vote soit utile non seulement aux millions de femmes que la loi protège en France mais aussi aux millions de celles dans le monde qu'aucune loi ne protège comme moi

merci beaucoup est à présent à Mme Mariole Battistel, pour le groupe socialiste de l'assemblée nationale.

Je ressens, avec une plénitude jamais connue à ce jour, accord entre ma fonction de législateur et ma condition de femme il nous appartient aujourd'hui de dire que l'ère du monde fini commence ces mots de gisèle halimi résonnent puissamment à sa tribune cet après midi et je l'ai fait bien il résonne d'autant plus fort pour moi qu'il aii l'honneur de représenter la quatrième circonscription de l'isère comme elle l'a fait en son temps et que ces combats ont influé les miens c'est ainsi avec une immense émotion honneur et fierté que je porte la voix des députés socialistes devant le parlement réunis en congrès en ce jour historique du quatre vingt un jour historique en ce qu'il est une victoire pour les femmes pour leurs droits si souvent discutés ballottés et mis à mal dépendant des changements politiques jamais à l'abri de les voir reculer c'est la victoire la victoire de simone de beauvoir qui nous appelait à la vigilance de notre vie durant

qui agissent au quotidien loin des dorures de nos tribunes pour que les lois et les grands principes soient des réalités concrètes qui protègent et libèrent les femmes dans la revendication et l'exercice de leur droit à disposer librement de leur corps, c'est notre victoire à toutes, oui face à ceux qui doutent encore que l'avortement mérite d'être défendu car comment fermer les yeux sur la décision des sept États américains ayant depuis l'arrêt de la Cour suprême interdit en cas de viol ou d'inceste, comment ne pas faire le parallèle quand certains de nos voisins européens comme la Pologne, la Hongrie, mais aussi le Portugal en conditionnent et en réduisent l'accès comment nee pas s'inquiéter que dans notre pays les entraves à l'ivg prennent des formes de pluss enplus, pernicieuses de la part des mouvements anti choix, jusque dans certains médias qui peut alors dans cette époque de doute et d'instabilité préjuger de ce qu'il pourrait advenir en france ainsi dans ce contexte global de remise en question du droit à l'avortement ce jour du quatre mars deux mille vingt quatre est historique aussi pour la france

parmi les valeurs intangibles et tout ce qui fait la force d'une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, la France perpétue l'inspiration a été son histoire constitutionnelle pour de nombreux pays, fidèle à son image humaniste. Notre nation s'érige en vigie des droits des femmes et montre le chemin Toutefois, si ce jour est historique, la constitutionnalisation, ce n'est pas une panthéon sation il ne s'agit pas de saluer un droit acquis et solide et de graver notre temple républicain aux grandes femmes. La patrie reconnaissante la constitutionnalisation telle que nous la réclamons, nous s socialistes, implique une réelle protection. Il ne s'agit pas uniquement d'inscrire notre droit mais bien de de nous donner les moyens de le rendre effectif. Il serait bien malvenu que tous de tous se réunir aujourd'hui pour consacrer un droit sans pour autant en garantir l'applicabilité. Ainsi, ce vote nous engage, pour les prochaines lois de financement de la sécurité sociale, à donner pluss de moyens à l'hôpital public, à la médecine de ville, à lutter contre les déserts médicaux, à renforcer le soutien public, aux associations, au planning familial, à la santé scolaire, pour accompagner toutes celles qui en ont besoin. En ce sens, nous aurions préféré voter plus ambitieux incluant la contraception mais nous savons que les victoires féministes ont toujours été le fruit de compromis dès lors que l'on en mille neuf cent soixante quinze l'opposition de gauche avait choisi la conviction plutôt que la posture pour faire adopter la loi veil ans plus tard nous continuons donc à adopter cette ligne constructive pour faire primer l'intérêt des femmes je veux ici saluer la responsabilité de la quasi totalité des forces politiques qui montrent que notre pays peut se rassembler dans le sens de l'histoire, parce qu'aujourd'hui, nous votons pour des milliers de femmes pour leurs droits, pour leur liberté, pour leur corps et pour leur vie, parce que par ce vote, nous contribuons à fonder une communauté politique, de citoyennes et de citoyens égaux parce que là où le droit est bien souvent en retard sur la société, il s'agit dès aujourd'hui de se prémunir Parce qu'il est de la responsabilité de la France, pays des droits humaine, d'envoyer un signal fort, qui transcende ses frontières. Les députés socialistes sont fiers de voter aujourd'hui pour graver l'inscription de l'ivg dans la norme suprême de la République. Je vous remercie

notre devise liberté, égalité, fraternité se font dans cette constitutionnalisation de l'ivg La liberté, d'abord, puisque ce texte permett à toutes les femmes de ce pays de disposer de leur corps librement, nous sommes libres de choisir ou non d'avoir un enfant et libres de choisir d'avorter gratuitement. L'égalité ensuite, puisque cette constitutionnalisation permet de lutter pour gommer la domination sur les femmes, c'est bien le travail du constituant d'œuvrer pour que ce principe d'égalité soit concret et protecteur. et enfin, la fraternité, puisque c'est l'unité qui anime ce texte réunissant le peuple français et l'humanité autour des valeurs de la République. La fraternité également en déstigmatiser les femmes qui ont recours à un avortement. Nous en sommes profondément convaincus. Le caractère solennel de ce moment m'invite à remercier toutes les femmes quii ont su lutter, au fil des siècles, pour ce droit et se défaire d'une société aliénante. Il est vrai que dans leur marche V. la liberté, les femmes ont toujours mené la lutte contre des forces réactionnaires et elles continuent de le faire aujourd'hui en France comme à l'étranger. Elles n'ont pas acquis leurs droits par la générosité du pouvoir, ils sont le résultat de cette lutte et, à quelques jours de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, je veux rappeler qu'il y en a encore tant d'autres à conquérir en france dans le monde notamment dans le domaine social et économique notre groupe notre sensibilité politique a toujours su se ranger du côté de ces femmes en mille

cette ambition est donc aujourd'hui une réalité c'est un moment important pour toutes les femmes sur le territoire français, mais c'est aussi un appel à tous les pays du monde à inscrire ce droit dans leur constitution s'il s'agit d'un combat fortement mené par les femmes, c'est surtout une avancée pour l'humanité tout entière d'une société dans son ensemble qui fait sien ce principe fondamental. Oui, les femmes ont le droit à disposer de leur corps, elles ont le droit à donner la la vie et à éduquer des enfants désirés et aimés, mais la maternité ne peut être imposée pour être réussie, la maternité doit être choisie partagée et non subi.

collègues, comme dans les territoires ruraux pour asseoir le droit concret à l'avortement le manque de moyens de l'hôpital public les nombreuses fermetures de centres v g de cent les difficultés à trouver des professionnels de santé disponibles et les déserts médicaux dans tout notre territoire placent de nombreuses femmes aujourd'hui dans notre pays dans une incapacité pratique d'exercer ce droit malheureusement les disparités territoriales ne sont pas que le reflet des politiques de santé publique dramatiques dans notre pays, et ce depuis plusieurs décennies, et la solennité vote d'aujourd'hui ne peut extraire les responsabilités politiques d'une situation au recul dans notre pays sur l'accès à ce droit. Il nous faudra donc continuer à lutter pour que toutes les femmes de tous les niveaux sociaux de tous les territoires aient effectivement accès à ce droit. Pour l'heure, nous saluons solennellement cette inscription dans la Constitution. le redis inscrire cette liberté individuelle La Constitution, c'est s'inscrire dans commun de liberté, d'égalité d'égalité et de fraternité. La République peut être fière et nous pouvons représentants du peuple français et de ces territoires être fiers de notre République. C'est bien pour réaffirmer que le droit à disposer de son corps est fondamental que le groupe communiste, républicain, citoyen écologiste kanakis votera pour ce projet de loi constitutionnel à présent à madame anne cécile violent pour le groupe horizon de l'assemblée nationale

Je remercie particulièrement mon président et mes collègues pour leur confiance. Voter ce projet de loi constitutionnel aujourd'hui dans cette salle de congrès, c'est envoyer un message historique aux femmes françaises. mais aussi aux femmes du monde entier Votre liberté de choisir fait partie intégrante des valeurs fondamentales de notre pays. Votre corps n'est pas un territoire à réguler, mais un espace de libre arbitre et d'autodétermination. Et je crois que nous pouvons en être fiers.

le 1ᵉʳ d'europe, le 1ᵉʳ dans le monde à protéger, au sein de sa constitution la santé physique et psychique des femmes contre les risques que présente un avortement dans la clandestinité. Oui, nous pouvons être fiers parce que cette constitutionnalisation et contrairement à ce qui a pu être dit, n'est pas qu'un symbole. elle est nécessaire et indispensable, la liberté de recourir à l'ivg nee fait l'objet actuellement d'aucune consécration dans nos textes fondateurs, nationaux ou européens et, si d'aventure elle était un jour menacée, il serait trop tard pour la protéger. Le Conseil d'état a été limpide sur ce point je le cite le caractère réversible et limité de la protection conférée par la loi ordinaire. justifie que soient garanties par la Constitution la liberté de la femme de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Soyons très clairs, tant mieux si cette liberté n'est jamais remise en cause, mais imaginez un peu si d'aventure nous nous retrouvions un jour dans une situation comparable aux états unis assumerez vous de dire à vos filles à vos pas soutenu à vos pas soutenu ce projet de loi constitutionnelle à l'époque simplement parce que je pensais que ça ne pourrait pas arriver chez nous alors même que certains de nos pays voisins. Européens remettent en cause cette liberté gouverner exige une Danti, ceci per les risques, c'est comme bâtir un rempart avant l'assaut, ne pas attendre la catastrophe pour se prémunir et en subir les conséquences néfastes. voilà la sagesse de l'assurance. Oui, nous pouvons être fiers parce que la rédaction qui nous est soumise aujourd'hui est le fruit d'un consensus transpartisane, dialogue entre deux chambres respectueux du travail de chacune et de chacun. de chacune et de chacun parce que oui, bien d'une histoire commune qui nous concerne. Les hommes comme les femmes et je tiens à vous remercier, M. le Garde des Sceaux, de vous être saisi de ce sujet avec tant de sincérité et d'engagement. Plus encore, elle me semble répondre point par point aux interrogations de chacun d'abord et, avant tout, elle protège la liberté d'abord et, avant tout, elle protège la liberté des femmes inscrite dans la Constitution. Le législateur ne pourra pas interdire tout recours à l'i Vg ni en restreindre les conditions d'exercice de façon telle qu'il priverait cette liberté de toute portée. Ensuite, elle ne consacre pas une garantie inconditionnelle de pouvoir recourir à l'ivg, comme droit ou liberté fondamentale. ou liberté fondamentale. Liberace a vocation à être conciliée avec d'autres droits fondamentaux que contiennent nos normes suprêmes, par exemple à ceux qui s'inquiètent de la création d'un éventuel déséquilibre entre deux principes à valeur constitutionnelle que sont la liberté de la femme et de la personne humaine contre toute forme de dégradation. Je réponds que ce n'est nullement le projet et l'intention de cette loi. Cette rédaction ne remet pas davantage en cause. la liberté constitutionnelle de conscience qui sous tend la liberté des médecins et des sages femmes de ne pas pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Enfin, cette rédaction affirme qu'il revient aux représentants du peuple de déterminer les conditions dans lesquelles cette liberté est exercée. Ainsi, la liberté de recourir à l'i Vg sera protégée de façon pérenne tout en continuant à être encadrée par un processus démocratique. Dans un contexte mondial où les attaques se multiplient contre l'accès à l'avortement, vous l'aurez compris, je crois profondément que ce projet de loi constitutionnelle doit être voté avec conviction. Détermination et fierté parce qu'ils consacrent la liberté de la femme la protection de ses choix, le rôle du peuple dans la fixation du cadre dans lequel s'exerce cette liberté Évidemment, le groupe horizon et apparenté votera en faveur de ce projet de loi, La parole est à Mᵐᵉ Mélanie Vogel, du groupe Écologie, Solidarité et Territoire du Sénat.

Par des femmes qui ont moins regardé pourquoi elle pouvait perdre que comment elle pouvaient gagner. gagner. il y a un an et demi quand j'ai proposé à mes collègues au sénat de mettre aux voix une proposition de loi transpartisane pour introduire le droit à l'i V G dans la Constitution, beaucoup m'ont dit oui. Mais tu sais, n'est ce pas que c'est impossible? jamais jamais le Sénat ne votera pour introduire le droit à l'i V G dans la Constitution la semaine dernière Encore, beaucoup pensaient que ce congrès était inaccessible, que le conservatisme serait plus fort et pourtant nous sommes là et c'est une magnifique leçon que nous nous donnons à nous mêmes. nous les féministes nous sommes si forts et si on ne lâche rien à la fin on gagne

la démonstration que nous avons faite avec mathilde panot avec aurore bergé avec laurence rossignol avec dominique verriez laurence cohen avec elsa chalk avec ses femmes qui ont choisi dans ce combat soixante quinze l'intérêt général par dessus toute autre considération c'est que la victoire ne pouvait être que soror et collective elle est celle de toutes celles et ceux qui se sont mobilisées célèbres connues ou anonymes, celles des militantes et des associations féministes qui n'ont jamais rien lâché, qui nous ont fait confiance, qui ont mobilisées sans répit. Merci, Bravo Celle de toutes ces personnes qui ont relayé nos appels, interpellé leurs élus, marché écrits, pris la parole, celles des femmes, des filles, des petites filles, des nièces de sénateurs, qui ont convaincu avec leurs mots, leur père, leur oncle, leurs maris, chacune chacun de vous qui à votre niveau avait agi soyez fiers de ce que nous avons fait ensemble le quatre mars deux mille vingt quatre est désormais gravé dans la grande histoire des droits humains et des droits des femmes comme un tournant historique alors que des siècles durant l'exercice par les femmes de leurs droits inhérents inhérents à la condition humaine de choisir leur vie alors que le simple exercice de ce droit leur a fait risquer la mort alors que pendant des siècles l'avortement caché secret tu un mot que l'on chuchotait la peur au ventre il s'inscrit aujourd'hui noir sur blanc au plus haut où nous pourrions l'inscrire dans la Constitution par cet acte d'une portée juridique et politique sans précédent. La République française reconnaît aujourd'hui, solennellement que le droit à l'avortement n'est plus une option, c'est une condition de notre démocratie qu'il n'y a pas. de société pleinement démocratique, libres et égalitaire. Quii ne s'interdisent d'interdire aux femmes de maîtriser leur destin, qu'ils n'aient pas de société pleinement démocratique, libre et égalitaire du droit des femmes à disposer de leur corps que la République française, désormais, ne sera plus jamais la République sans le droit à l'avortement. C'est un message Pour toutes les Françaises et les Français qui tiennent tant à ce droit et réclamaient massivement dans la Constitution un message pour toutes celles qui ont connu le temps où le prix du choix pouvait être l'exclusion la prison ou la mort qui ont connu l'humiliation de la clandestinité la douleur des curetage sans anesthésie les cintres et les aiguilles un message à celles qui ont pleuré de joie de soulagement le dix sept janvier mille jamais vos filles vos petites filles vos nièces ne connaîtront cela sommes à jamais libres vous avez définitivement gagné

sans trembler cet horizon a disparu Vous avez définitivement perdu, plus jamais nous ne reviendrons sur le droit à l'i V. G. G. C'est aussi un message pour le monde entier, un message aux Américaines, aux Argentines, aux Hongroises, aux Polonaises, aux Allemandes, aux Iraniennes et aux Marocaines, à toutes celles qui, dans le monde, vivent toujours ou de ou de nouveau le martyre des cintres, la douleur des tricoteuses, l'angoisse la peur de la prison et le risque de la mort à toutes celles qui craignent de les revivre, à toutes celles qui se battent pour acquérir, conserver ou élargir leurs nous sommes inconditionnellement avec vous, le recul des droits sexuels et reproductifs dans le monde, n'est pas une fatalité, vous pouvez gagner, nous pouvons gagner, car ensembles unis et solidaires, notre pouvoir est sans limite, nous pouvons renvoyer le patriarcat, l'obscurantisme religieux, la domination masculine dans le cimetière des idées réactionnaires nous sommes si forts et si le pire n'est jamais incertain le meilleur lui est toujours possible possible qui semble perdu d'avance, c'est notre victoire de demain je vous remercie, La parole est à Mᵐᵉ la présidente Cyril Chatelin, pour le groupe écologiste de l'assemblée nationale

utérus transpercés, dans le vagin des utérus transpercés, des cintres enfoncés, les infections de Javel, des sondes qui restent dans le corps un deux, trois jours, des curetage à vif, des hémorragies, des septicémies la mémoire des femmes qu'on a traînées devant les tribunaux les sans argent sans relation les pluss vulnérables la mémoire de la colère le torchon brûle la gerbe pour la femme du soldat inconnu le manifeste des trois cent quarante trois la plaidoirie de gie halimi et le discours de simone veil aujourd'hui nous nous tenons sur l'épaule des géantes nous faisons partie d'une chaîne invisible les femmes quii avortent les faiseuses d'anges les porteuses millénaires, les femmes épuisées par des grossesses non désirées, les femmes qui, par leur parole ou par leur silence, ont transmis à leurs filles, la certitude que jamais elles ne céderaient et elle ne se soumettraient à la loi des hommes, les femmes qui ont posé les mots, les femmes qui ont raconté les femmes qui n'ont pas pu, qui n'ont pas voulu le dire car elles l'ont gardé comme un secret, parfois comme une honte car cela ne se faisait pas, cela ne se disait pas les femmes qui en sont mortes, les femmes qui ont donné des adresses et les femmes qui ont organisé l'écart pour l'étranger. Carl Long est notre lutte, nous nous sommes reconnus, nous nous sommes découvertes des milliers et des millions et nous partageons un même combat, un combat qui se transmet de mère en fille, d'amis en confidente, d'inconnus inconnus une force qui s'est transformée en mouvement, la maternité heureuse, le mouvement français pour le planning familial, le mouvement de libération des femmes, le mouvement pour la liberté, de l'avortement et de la contraception des mouvements qui se sont transformés en raz de marée, une déferlante, contre un dogme que le corps des femmes ne leur appartenait pas, qu'il a un pas qu'il appartenait à leurs pères, à leurs maris ou à la nation, un dogme longtemps assenés par la loi, par la religion, un dogme qui est encore tenace, celui des corps féminins

neuf cent soixante quinze en france l'avortement enfin est légal mais il n'existait pas jusqu'au vote qui nous réunit de protection de la liberté et de l'interruption volontaire de grossesse par le juge constitutionnel ce que la loi a pu faire la loi pouvait le défaire douze lorsque s'ouvre le procès de bobigny nous sommes dans la cinquième république nous avons la même constitution qu'aujourd'hui et et les femmes qui avortent et toutes ceux et toutes celles qui leur viennent en aide sont traitées comme des criminels nous nous parlementaires ici réunis nous reconnaissons l'interruption volontaire de grossesse comme une liberté fondamentale de la même importance que l'ensemble des droits et des libertés garanties par notre Constitution, nous réaffirmons le rôle du Parlement afin d'établir les conditions d'exercice et de les garantir. Car, pour qu'une liberté s'exerce, elle doit être concrètement possible et cela reste encore trop difficile car les temps d'attente sont trop longs, les praticiens trop peu nombreux, l'éducation à la vie affective et sexuelle encore balbutiante le travail parlementaire va continuer. Oui, le combat féministe n'est pas terminé mais aujourd'hui, savourons cette loi qui marque un nouveau jalon dans l'histoire de France, une nouvelle conquête dans la lutte des femmes, une conquête pour laquelle je tiens à remercier les militantes féministes qui ont marché, qui ont fait signer des pétitions qui ont tenu des stands dans toute la France pour dire nous devons faire entrer l'i V G dans la Constitution. Cette constitutionnalisation de l'i V G. c'est votre victoire. à saluer le travail essentiel de quatre parlementaires Mélanie Veule, sénatrice écologiste, Mathilde Panot, députée présidente du groupe La France insoumise, Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, est Aurore Bergé, alors députée et présidente du groupe. Ensemble, elles nous ont conduits à ce vote un pari qui pouvait sembler fou pour qui nee connaîtrait pas la puissance d'une idée dont le temps est venu. À mes filles, à toutes les femmes de France, à toutes celles qui se poseront la question est ce que je peux le garder, est ce que je veux le garder, nous parlementaires, nous vous le garantissons nul? Nee peut vous contraindre, nul ne peut vous forcer, nul nee peut vous intimider, null nee peut vous intimider, vous obliger, vous êtes les maîtresses de votre destinée. Notre cœur, nos choix?

La parole est à Mᵐᵉ la présidente Maryse Carrère, pour le groupe Rassemblement démocratique social européen du Sénat.

Mᵐᵉ la Présidente du Congrès, M. le Président du Sénat, M. le 1ᵉʳ ministre, M. le Garde des Sceaux, Mᵐᵉˢ et MM. les ministres, mes chers collègues, il aura fallu trois textes avant que soit enfin soumise au Congrès la possibilité d'inscrire dans la Constitution la liberté de recourir à l'Cerruti, volontaire de grossesse. Et je salue le la détermination de tous nos collègues qui ont porté ce combat, en particulier du côté du Sénat, les sénatrices Mélanie Vaugelas, Vogel, Laurence Rossignol, Laurence Cohen, Mélanie Dominique, Veria Pardon et bien d'autres, ainsi que toutes les personnalités qui sont venues en renfort à ce v. leur prise de position publique. Merci aussi M. le garde des sceaux d'avoir concrétisé ces espoirs. Je salue également la bienveillance de la commission des lois du Sénat et qui méritent d'être soulignées car sa majorité a su laisser de côté ses quelques réserves pour rechercher le compromis dans l'intérêt d'une liberté chère aux femmes. Plus largement, mercredi dernier, le Sénat a été au rendez vous du pacte républicain dont les valeurs fondatrices nous invitent, autant que nécessaire, à ériger des digues autour des droits fondamentaux Rappelons qu'au cours de l'examen de la loi Veil, la chambre haute avait porté plusieurs mesures progressistes dont le remboursement de l'ivg j'ajouterai que les sénateurs avaient très largement adopté le texte rapporté à l'époque par jean mézard aujourd'hui pourquoi tant de précautions bientôt cinquantenaire la loi de soixante quinze par sa longévité nee démontre t elle pas sa résistance et la réponse est dans les proposs de simone de beauvoir et vous l'avez rappelé monsieur le premier ministre n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique économique ou religieuses pour que les droits des femmes soient remis en question. Entre régime autoritaire et progression des populismes dans les démocraties, même dans les plus grandes, on observe un recul des libertés d'un bout à l'autre de la planète bien souvent les femmes sont les premières victimes de ces reculs et les plus modestes avant les des autres c'est le cas outre atlantique depuis que la cour suprême américaine a révoqué en deux mille vingt deux la protection au niveau fédéral du droit à l'avortement c'est le cas dans plusieurs pays de l'union européenne où les conditions de l'accès à l'ivg ont été durcies en france qui peut prétendre que le mouvement pro vi ne trouverait pas son audience si demain le contexte venait à changer radicalement. De surcroît, si par dessus certains médias venaient à l'appuyer, comme on a pu le déplorer récemment avec la diffusion par une chaîne privée d'une infographie nauséabonde, simple négligence ou véritable complaisance. Nous avons bien entendu les excuses, mais Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas naïfs et, face à tout cela, nous devons opposera vigilance aussi le D S E approuve à l'unanimité l'inscription de l'i V G dans la constitution, malgré cette nécessité évidente. Certains mettent en doute la solidité d'une constitutionnalisation qui ne serait qu'illusoire et symbolique parce qu'elle ne résoudrait pas les problèmes d'accès à l'ivg C'est au législateur et au pouvoir réglementaire qu'il revient de créer les conditions de l'accès à tous les droits inscrits dans la constitution, il va de soi que mon groupe sera attentif aux conditions matérielles de l'accès à l'ivg à l'i V G sur tous les territoires ainsi qu'à l'effectivité des politiques de prévention, ceci étant dit notre Constitution doit afficher des principes, des valeurs et des objectifs elle indique la finalité de notre droit celle à laquelle il ne saurait déroger de toute évidence la garantie donnée à la liberté des femmes d'interrompre leur grossesse trouvera sa place dans un tel corpus en particulier à l'article trente quatre chacun a ses convictions religieuses idéologiques celles ci ne sauraient être retranchées derrière le droit faute d'être clairement assumé pour le d s e je le répète il n'y a aucun doute nous souhaitons écarter le risque de voir l'i V G aux prises avec un conservatisme conquérant ou des fanatismes religieux, au nom de la laïcité notre République doit mettre à l'abri des droits sociaux du mieux qu'elle peut enfin. il est coutume de dire que la défense de l'i V G est un combat de femmes pour les femmes. Oui, à l'évidence mais le dramatique chemin qui mène V. l'i V G a forcément commencé à deux, dans certains cas, c'est également la liberté des hommes qui est engagée C'est pourquoi mes chers collègues nous avons aujourd'hui l'immense responsabilité collective de le sanctuariser nous le devons à toutes celles et à tous ceux qui se sont battus pour cet dépénalisation il y a cinquante

La parole est à Mᵐᵉ Elsa Foncillon, pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Mᵐᵉ la Présidente, M. le Président, M. le 1ᵉʳ ministre, M. le Garde des Sceaux. Chers collègues, c'est avec une grande émotion, mais aussi disons le un grand bonheur que j'interviens aujourd'hui au nom du groupe d pour ce vote si important pour notre pays et si décisif dans la vie des femmes ce matin l'une des signataires du manifeste des s'adressaient ainsi aux jeunes femmes elle leur disait vous avez dépassé nos rêves on n'a jamais imaginé que le droit à l'i v g pourrait être inscrit dans la constitution alors madame à notre tour de vous dire merci merci à vous à toutes celles qui nous ont menés sursangle min car sans vos luttes rien de tout cela n'aurait été possible. je veux dire aussi merci à ces femmes, nièces, filles ou petites filles de parlementaires qui ont contribué au vote décisif du En En ce jour, avec les députés de mon groupe, nous adressons toute notre solidarité, tout notre soutien, notre force aussi aux femmes qui défendent ce droit à travers le pour cela harcèlement, stigmatisation, violences physiques aussi et des procès. Je crois que les régressions, comme les conquêtes, ont une résonance mondiale. Alors force à vous, Mᵐᵉˢ Nous pensons également à ces femmes obligées d'écouter le corps du fœtus parce qu'une loi les yy oblige à celles qui mettent toutes leurs économies dans un déplacement vers un autre pays pour pouvoir avorter quarante sept par an dans le monde qui meurent encore d'un avortement clandestin parce que chers collègues les femmes qui veulent avorter avortent c'est le cas depuis la nuit des temps lorsqu'elles n'ont pas ce droit elles trouvent tous les moyens possibles pour mettre fin à cette grossesse y compris quitte à mettre vie en péril. Cette constitutionnalisation est loin, pour nous, de n'être qu'un symbole Nous savons que, même dans les grandes démocraties, le retour en arrière est possible, nous savons aussi que, lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir, elle s'en prend d'abord aux droits des femmes et particulièrement à leurs droits reproductifs. Alors à ceux qui nous ont expliqué que ce droit n'était ici pas en danger, je veux leur dire qu'il suffit de regarder la vigueur et l'indignité aussi, avec lesquels les anti choix et les gardiens du Patriarcat ont redoublé d'efforts pour que ce vote, ici au Congrès n'a advienne pas à ceux qui nous ont adressé des fœtus en plastique des fascicules faisant parler les embryons qui ont comparé l'avortement à un meurtre. Sachez que vous avez décuplé la force des féministes, sachez que vous avez perdu perdu Pour nos mères, nos filles et nos sœurs, d'ici et d'ailleurs, nous affirmons maintenant et ici que le droit à disposer de son corps est un droit fondamental et il est essentiel à la liberté individuelle. Il est donc une condition indispensable à l'existence de toutes les autres libertés liberté, égalité, sauroit. aussi pour nous une manière de se prémunir de ces politiques nationalistes qui font du ventre des femmes des femmes une variable d'ajustement démographique, au mépris des droits fondamentaux.

pour différentes raisons d'abord parce que les des conditions à ce droit peuvent être ajoutées et malheureusement pour le pire ensuite parce qu'il ne prend pas en compte le droit à la contraception quii est pourtant la cible privilégiée des attaques de ceux qui veulent s'attaquer au droit à l'iv ces compromis nous les avons faits pour aboutir, nous les assumons et nous en sommes fiers à l'issue qui se profile. Mais sachez que nous ne lâchons jamais parce que nos corps nous appartiennent et nos choix aussi

les personnes en situation de pauvreté, de migration d'exclusion et les personnes mineures en sont les premières victimes lors du procès de bobigny gisèle halimi nous avertissait elle disait c'est toujours la même classe celle des femmes pauvres vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans argent et sans relations quii est frappée. Alors, ce vote nous engage, vous engage, Mᵐᵉˢ et MM. les ministres à garantir ce droit aussi par des moyens dans ce domaine. Enfin, j'espère que ce vote participera ou contribuera à lever le tabou qui règne encore sur l'avortement, permettant ainsi de ne pas culpabiliser celles pour qui ce n'est pas un drame d'avorter et permettant à celles pour lesquelles la décision ou le chemin sont plus difficiles de trouver les appuis nécessaires. Pour finir, parce que nous ne savons que trop bien que ce vote historique aujourd'hui entraînera aussi, dès demain, son lot, de son lot de contre offensives réactionnaires. Eh bien, rendez vous dès demain et nombreux, le 8 mars pour la grève féministe, pour de nouvelles conquêtes féministes, pour l'égalité salariale et pour que nos luttes se transforment en victoire, merci beaucoup ma chère collègue la parole est à monsieur le président bertrand pancher pour le groupe liberté indépendant outre mer et territoire de l'assemblée nationale la nationale la présidente du congrès monsieur le président du sénat monsieur le premier ministre messieurs les ministres chers collègues sénateurs et députés étant le dernier orateur, merci pour votre patience. La lutte pour les droits des femmes et pour l'égalité entre les hommes et les femmes est un long chemin. Et elle a subi tellement de recul Hongrie, Pologne, États Unis, Argentine, sans parler de la situation dramatique des femmes en Afghanistan ou Iran. Femmes vit liberté réprimée dans le sang et je veux avoir à cette tribune au nom des collègues du groupe Iot une pensée toute particulière pour les femmes qui souffrent dans le monde du simple fait qu'elles sont des femmes ou parce qu'elles luttent pour leurs droits. Cette lutte connaît chez nous, aujourd'hui, maintenant deux avancées. la 1ʳᵉ, c'est de voir ce Congrès présidé pour la 1ʳᵉ fois par une femme. La 2ᵈᵉ est évidemment l'inscription de la liberté garantie de recourir à l'i V G. dans notre Constitution. Là encore, je pense à toutes les femmes qui, par le passé, ont été condamnées pour avoir eu recours à l'avortement, qui ont eu à connaître clandestinité, au propre des honneurs, c'est pour y mettre fin que Simone Veil mena, il y a 50 ans combat pour légaliser l'accès à l'ivg nous avons tous en mémoire la violence des débats, les attaques dont elle fut la cible et les affronta avec un courage et une détermination sans faille. Il nous faut nous réjouir que les débats, aujourd'hui, comme lors de l'examen des textes, tant à l'assemblée qu'au Sénat, ait se soient tenus dans une atmosphère globalement apaisée. Au final, nous avons à voter un texte de compromis qui consacre la liberté garantie aux femmes de recourir à l'ivg, la liberté de choisir et de disposer de leur corps. Les membres de mon groupe se prononceront comme toujours à la lumière de ce que dicte leur conscience mais très très majoritairement en faveur de ce texte. J'entends les arguments de ceux pour qui cette réforme est superflue. J'entends aussi les réserves exprimées J'entends aussi celle ceux qui, parmi nos concitoyens, nous disent qu'il y a tant d'autres priorités la crise agricole, la vie chère, la guerre en Ukraine, l'état de nos services publics. ne remet ce droit en cause aujourd'hui mais quand sera t il demain? Nous avons tous cette citation de Beauvoir en tête Il suffira d'une crise politique, économique et religieuse pour que le droit des femmes soient remis en question. Aujourd'hui, nous gravons cette liberté dans la norme suprême, nous lui donnons plus de force et ce vote s'inscrit dans le prolongement du combat universaliste et humaniste de la France. Cette consécration constitutionnelle ne marque pourtant pas la fin des combats pour les femmes. Je pense aux combats pour l'égalité tant qu'il reste à faire pour l'égalité professionnelle et économique où persiste trop souvent le plafond de verre des salaires pour lutter contre les violences faites aux femmes et féminicides ou encore sur la question de la santé des femmes pour autant grande cause du quinquennat depuis deux mille dix sept les progrès restent trop lents ce vote nee marque pas non plus la fin du combat pour le droit effectif de l'ivg dans notre pays trop souvent les femmes rencontrent des obstacles difficultés d'accès à l'information à des praticiens, délais d'intervention trop long. Comme dans de nombreux domaines, les fractures sociales, pour elles, se cumulent aux fractures territoriales est donc tout aussi important de proclamer une liberté que de mettre en œuvre les conditions d'exercice de cette liberté. de santé publique, moyens alloués à nos politiques de santé publique, à la prévention, à l'éducation sexuelle et à la contraception chez les jeunes comme dans d'autres pays qui l'ont fait. Je pense notamment à l'exemple remarquable des pays bas

et puisque nous sommes réunis pour modifier notre constitution comment ne pas aussi chers collègues députés et sénateurs exiger des réformes d'ampleur institutionnelle pour résoudre notamment la démocratique que nous traversons afin d'éviter que les extrémistes arrivent au pouvoir et remettent tout en cause. le seul pays où tout se décide au niveau central, mais comment voulez vous que cela marche, un pays qui se meurt dans une gouvernance verticale jupitérienne? d'une Sud minist Ation étouffante, le seul pays qui ne donne jamais la parole aux peuple, l'adaptation législative et réglementaire aux territoires qui le réclament pour tout ce qui est non régalien, doit être consacré, tout comme la généralisation des référendums et le renforcement du rôle du Parlement. le seul pays où l'on ne fait pas confiance au corps intermédiaire, aux partenaires sociaux pour gérer la protection du chômage, de la protection sociale, des retraites complémentaires, Agir Arco Assurance chômage. oui nous saluons l'inscription de l'ivg dans notre constitution nous nous en réjouissons mais il y a encore, chers collègues, tant et tant de chemin à faire. de chemin à faire. M. le Président, merci beaucoup, nous avons les explications de vote je vais maintenant mettre aux voix le projet de loi constitutionnel relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse

Mes chers collègues, la séance est reprise. voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnel nombre de votants neuf cents deux nombre de suffrages exprimés huit

douze merci pour elle le congrès a adopté le projet de loi constitutionnel relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse approuvée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés sera transmis à m le président de la république je vous remercie la séance est levée

Merci